il n'y a pas forcément de lien entre le régime dont dépend l'entreprise et l'importance ou non de la pollution du sol qu'elle peut engendrer.

contrôlée par l'administration, peut avoir pollué les sols de manière beaucoup plus significative qu'une ICPE autorisée ou enregistrée. Cet amendement tend à rétablir une égalité de traitement dans les mesures de gestion des sites pollués.

des mesures de réhabilitation ainsi que la mise en oeuvre des mesures de mise en sécurité des sites. Or l'appréciation de la pertinence des mesures ressortit à la seule autorité compétente ayant autorisé le projet, ces mesures faisant l'objet d'une décision administrative. En aucun cas, les prescriptions de réhabilitation ni même de mise en sécurité ne doivent être transférées à une entreprise tierce, même certifiée, dont les actes sont insusceptibles de recours. En outre, la mise en sécurité participant en tant que telle à la réhabilitation d'un site, il n'y a pas lieu de dissocier ces deux opérations.

et de leur application. Cette disposition est utile, mais l'article crée une disparité de traitement selon le régime ICPE. Ainsi, si les installations soumises à autorisation et à enregistrement doivent faire attester de la mise en sécurité et de la réhabilitation,

car l'état de pollution lié à une activité ne dépend pas de son régime ICPE. Une installation soumise à déclaration, qui a pu être moins contrôlée par l'administration, peut très bien avoir pollué le site au même titre qu'une ICPE autorisée ou enregistrée. Cet amendement vise ainsi à ce que les installations soumises à déclaration doivent également faire attester par un bureau d'études spécialisé indépendant de la mise en oeuvre des mesures de réhabilitation, et pas seulement de la mise en sécurité du site. Il ne faut néanmoins pas oublier que l'attestation des mesures prises semble être de la compétence des services déconcentrés de l'État. S'il est plus prudent d'exiger une telle attestation

? L'amendement n° 71 vise à étendre aux ICPE soumises à déclaration l'attestation par une entreprise certifiée de la pertinence et de la mise en oeuvre des mesures de réhabilitation du site après mise à l'arrêt, en complément des mesures de mise en sécurité déjà mentionnées dans le projet de loi initial. L'obligation d'avoir recours à une entreprise certifiée doit être ciblée sur les installations qui présentent des enjeux significatifs en termes de dépollution.

la mise en sécurité et la remise en état sont bien deux exercices distincts, qu'il convient de mentionner. En outre, il nous paraît important que l'entreprise certifiée examine la pertinence des mesures proposées afin d'assurer à l'inspection, sans préjudice de ses pouvoirs de police, qui demeurent inchangés, que ces opérations ont été réalisées comme attendu. L'intervention de ce tiers qualifié permettra de fiabiliser les mesures de dépollution.

le code de l'environnement distingue bien, au niveau réglementaire, deux opérations successives dans le processus de cessation d'activité d'une ICPE : la mise en sécurité, puis la réhabilitation ou la remise en état du site. L'objet de l'article 27 du projet de loi est de permettre l'attestation par un tiers certifié de la bonne mise en oeuvre de ces deux opérations, afin d'assurer à l'inspection des installations classées, sans préjudice de ses pouvoirs de police, qui demeurent inchangés, que ces opérations ont été réalisées conformément à l'attendu. Concrètement, pour les installations soumises à autorisation et à enregistrement, le mémoire de réhabilitation fera l'objet d'une première validation par une entreprise certifiée distincte de l'exploitant, qui pourra ainsi s'assurer du respect de la méthodologie appliquée, y compris pour les éventuels prélèvements destinés à caractériser la pollution. Bien entendu, l'inspection ne perd aucunement la possibilité de prescrire des mesures supplémentaires ou de préciser les objectifs à atteindre. en fait, d'une bonne répartition du travail. Enfin, les dispositions de cet article ne viendront pas remettre en cause le pouvoir de police du préfet et de l'inspection des installations classées, qui pourront toujours intervenir, même après la remise en état, pour prescrire les mesures nécessaires à la protection de l'environnement. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable

L'automatisation de la coordination entre la prorogation du permis de construire et celle de l'enquête publique associée relève de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Elle est en cours de rédaction par le ministère de la cohésion des territoires. Cette demande sera donc satisfaite dans les prochains mois.

à son fournisseur d'énergie le soin de conclure pour son compte un contrat d'accès au réseau, soit choisir de contractualiser lui-même. Pour garantir à tous les utilisateurs les mêmes droits d'accès au réseau, quel que soit leur choix, une uniformisation serait bénéfique et permettrait une gestion

Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, l'enfer de l'industrie grosse consommatrice en déborde, car ce ne sont pas les colloques, les missions, les articles, les déclarations qui font défaut : tout le monde soutient notre industrie grosse consommatrice et personne n'imagine qu'on ne la soutienne

à travers la mobilisation de l'hydraulique. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai souvenir d'une déclaration d'un des grands patrons de Péchiney dont le seul regret, à l'époque, était de n'avoir pu mobiliser l'hydraulique au fil de l'eau pour pouvoir soutenir l'aluminium français.

Ces difficultés sont d'autant plus grandes et incompréhensibles que ces industriels ont fait des efforts considérables et qu'ils sont prêts à se mobiliser sur des modes

Le soutien aux entreprises électro-intensives, tel que le promeuvent les auteurs de cet amendement, est essentiel pour notre compétitivité. Ces entreprises, très présentes dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie, de la papeterie et de la cimenterie, concentrent les deux tiers de la consommation électrique industrielle. Dans ces conditions, un contrat spécifique entre ces consommateurs et leurs fournisseurs, leur permettant un approvisionnement sur le long terme, est tout à fait intéressant. Pour autant, un tel dispositif pose des enjeux en termes de liberté contractuelle et emporte des conséquences juridiques et financières sur les fournisseurs d'électricité qu'il est nécessaire de bien mesurer avant d'envisager une évolution législative. Dans ce contexte, je vous propose de suivre l'avis du Gouvernement.

Le Gouvernement travaille donc à une nouvelle régulation économique du nucléaire existant, conformément au droit européen, et bénéficiant à tous les consommateurs au travers de l'Arenh 2. Je partage totalement l'objectif de

L'objet de l'amendement est simplificateur, puisqu'il s'agit de permettre à un gestionnaire de réseau de transport d'électricité de réaliser ou de faire réaliser, à la demande d'un producteur et à ses frais, des travaux de pose de fibre optique. Cependant, cette évolution interroge les missions des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, emporte des implications juridiques et financières entre ces derniers et les producteurs et soulève également des enjeux en termes de respect du droit de de la concurrence. Dans ces conditions, et eu égard à la technicité de la matière, il me semble préférable de suivre ici encore l'avis du Gouvernement.

afin de déterminer, par exemple, le montant des dotations versées par l'État ou tout simplement l'effectif des conseils municipaux. Il est possible de sanctionner tout refus de répondre à ce recensement par une amende de 38 euros,

cas échéant, le président de l'EPCI devant saisir le tribunal de police pour demander une sanction à l'encontre de la personne qui ne répond pas- et cela pour amende de 38 euros ... Dans le même esprit que ce projet de loi, cet amendement vise à faciliter les opérations d'enquête de recensement menées par les collectivités locales en leur permettant de solliciter auprès d'un fournisseur de biens ou de services la communication des informations nécessaires la communication des informations nécessaires à ces opérations de recensement en cas de défaut de réponse de l'administré concerné et après- j'y insiste -mise en demeure restée vaine. Quel Cet amendement pose plusieurs problèmes. Sur la forme, il tend à modifier l'article 7 de la loi de 1951.

la proportionnalité de la mesure au regard de l'ingérence dans la vie privée des particuliers est douteuse. D'ailleurs, en application de la loi de 1978 et du RGPD, chaque mairie devra faire une analyse d'impact,

d'indépendance selon lequel les statistiques sont développées, produites, diffusées d'une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser,

Je propose donc de changer cette situation par une double action législative : d'une part, publier chaque année la liste des procédures soumises à dérogation en vertu des principes généraux ; d'autre part, supprimer la possibilité pour le Gouvernement d'écarter les procédures de bonne administration.

Une partition claire est aujourd'hui indispensable. Si les exceptions deviennent la règle, il n'existe plus de principe général. Je partage pleinement le constat dressé par les auteurs de cet amendement : l'application de ce principe fonctionne mal. Toutefois, le dispositif proposé ne semble pas encore suffisamment abouti et complet pour apporter une vraie réponse.

les possibilités de dérogation strictement encadrées par l'article L. 231-5- nécessité de motifs de fond tenant à l'objet de la décision ou à la bonne administration et obligation procédurale de passer par un décret en conseil des ministres et en Conseil d'État

hors des cas actuellement visés par l'article L. 231-4. La liste mentionnée par le nouvel alinéa proposé semble se présenter comme le détail des dérogations permises par les alinéas précédents, qui ne mentionnent pas les motifs liés à l'objet des décisions et à la bonne administration. Il en résulte qu'il ne serait plus possible de déroger à la règle pour de tels motifs, ce qui nous paraît vraiment très inopportun. En outre, les dérogations qui existent actuellement deviendraient caduques, faute de base légale. Si la liste envisagée devait être comprise comme complétant les dérogations permises par les alinéas précédant l'article L. 231-4, 231-4, la rédaction proposée ne permettrait pas de s'assurer que le législateur prendrait la main sur cette liste, ainsi que l'affirme l'exposé des motifs, puisque l'amendement n'identifie ni l'auteur de cette liste ni ses modalités de publication, renvoyées à un décret simple.

? Cet amendement tend à introduire une déclaration d'établissement pour tout nouveau résident d'une commune. L'intention des auteurs de l'amendement est compréhensible : les maires peuvent parfois regretter de ne disposer que d'une information parcellaire

Deuxièmement, il semble paradoxal de prévoir, dans un projet de loi censé répondre à un besoin de simplification de l'action publique, une procédure administrative relativement lourde. Cette pesanteur administrative porterait sur les citoyens, mais également sur les maires

-du désaccord profond de notre groupe sur la manière dont l'article 45 de la Constitution a été appliqué à ce texte. Comme chacun le sait, cet article prévoit que tout amendement est recevable dès lors qu'il présente un rapport, même indirect, avec le texte

L'inscription aux registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile conditionne l'obtention de la reconnaissance et du bénéfice du statut de personnel navigant. Ce statut permet notamment de bénéficier du régime de protection sociale et de retraite complémentaire de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Le statut de personnel navigant est conditionné à l'exercice de l'une des quatre catégories de fonction énumérées par l'article L. 6521-1 du code des transports

Cet article supprime ces quatre catégories. L'obtention du statut de navigant professionnel de l'aéronautique civile dépendrait désormais de deux conditions exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ; deuxièmement, être titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ou relever des règlements européens applicables au personnel navigant. Nous nous interrogeons sur le nouveau périmètre du statut de personnel navigant. Les personnels qui exercent l'une des quatre catégories de fonction précédemment énumérées auront-ils toujours le droit

de surcroît aucun droit au personnel navigant. Ainsi, l'affiliation au régime de retraite des personnels navigants n'est aujourd'hui en aucun cas conditionnée à l'inscription au registre.

de nouvelles professions créées par la réglementation européenne. Par exemple, les membres d'équipage technique, les TCM, en secours médical d'urgence héliporté ne sont pas pris en compte par les registres.

répond davantage au droit canon de la libéralisation et de la concurrence, parfois érigé en dogme, plutôt qu'à la volonté de proximité, de présence territoriale et de maillage que vous prétendez afficher dans ce projet de loi de loi ? Ne sommes-nous pas aux antipodes des conclusions du grand débat, dont ce projet de loi est l'une des conclusions ? Où est la proximité ? Où est le maillage ? Où est l'écoute ? Finalement, ne faites-vous pas vôtre cette nouvelle maxime de l'action gouvernementale les gilets jaunes n'y pensaient pas, le Gouvernement l'a fait quand même

Les modalités de transmission des informations relatives à cette activité doivent pouvoir être modifiées afin de sécuriser le nombre de pharmaciens adjoints et de simplifier le travail des inspecteurs de chaque agence régionale de santé. Les précisions apportées à l'article L. 5125-33 du code de la santé publique sécurisent l'activité de vente en ligne en renforçant le rôle du pharmacien titulaire de l'officine, garantissant ainsi la sécurité et la traçabilité des médicaments.

Il s'agit bien d'une simplification, car nous proposons de mettre en place un régime de déclaration, et non d'autorisation, tout en permettant aux agences régionales de santé un meilleur contrôle. Nous voulons aussi faire évoluer les règles fixant le nombre de pharmaciens adjoints à recruter pour garantir la sécurité, la dispensation des produits ou encore la réalisation du conseil pharmaceutique. S'agissant de la vente de médicaments en ligne, elle est déjà autorisée- il n'y a aucune ambiguïté sur ce sur ce point -, et elle est nécessairement reliée à l'exercice du métier de pharmacien. C'est donc très exactement le contraire de ce qui a pu être indiqué. Il n'a jamais été question, y compris dans la rédaction initiale, de séparer le métier de pharmacien

point. En l'occurrence, le présent amendement vise à simplifier le cadre juridique relatif à la vente en ligne de médicaments, en passant d'un régime

rectifié. Faut-il rappeler la genèse de l'article 34, qui visait, il y a encore quelques jours, à développer des plateformes de vente en ligne de médicaments et, dans un but de compétitivité, à réduire le nombre de professionnels au sein des officines ?

Enfin, la mise en oeuvre de vos propositions se serait faite au détriment du maillage territorial constitué par les pharmaciens et, donc, au détriment de la demande de proximité exprimée par les Français.

comme Amazon. Nous avons rencontré les syndicats de pharmaciens et, dans l'attente du texte de concertation avec les professionnels, notre groupe a proposé la suppression de l'article en commission. alors prématuré de proposer une nouvelle rédaction de l'article. La concertation ayant finalement abouti, nous présentons cet amendement, qui reprend les objectifs de simplification tout en rappelant l'importance de l'expertise du pharmacien dans l'acte de vente d'un médicament, qui n'est pas une vente comme une autre. La profession a beaucoup oeuvré pour faire évoluer son activité, et cet amendement est aussi une reconnaissance de la coconstruction des règles. En matière de simplification, l'amendement permettra le passage au régime de déclaration, et non plus d'autorisation, pour l'activité

et qui a été travaillé avec les pharmaciens d'officine, vise à préciser le dispositif de l'article 34 du projet de loi. La pharmacie d'officine est un espace réglementé. La globalité de son activité doit être prise en compte pour déterminer le nombre de pharmaciens adjoints. Les modalités de transmission des informations relatives à cette activité doivent pouvoir être modifiées afin de sécuriser le nombre de pharmaciens adjoints et de simplifier le travail des inspecteurs de chaque agence régionale de santé.

Quant aux modalités de vente en ligne, on ne peut que se réjouir de l'abandon des notions de plateformes et de local détaché, qui présentaient un risque réel de remodelage, non seulement du paysage officinal, mais également de la sécurité de la dispensation.

alors qu'actuellement toute décision de l'ARS relative à la couverture des zones potentiellement atteintes par une pénurie de médicaments doit être prise dans le cadre d'une convention avec avec les représentants de la profession. Par ailleurs, l'inscription dans la loi d'un critère démographique de 1 500 habitants ne me paraît pas opportune pour apprécier la sous-densité d'une zone.

Ainsi, lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle autorisation peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert ou de regroupement dans cette commune.

le domicile est distingué de la résidence, qui est définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d'une manière assez stable, sans qu'elle constitue toujours son domicile. La notion de résidence que le que le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles préfèrent parfois à celle de domicile a pour principal enjeu d'inclure au sein des personnes éligibles à certaines prestations des personnes dépourvues de domicile stable. stable. Ainsi, l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, « pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile

en obtention de droits de la part de particuliers. L'amendement vise à renforcer la conditionnalité du versement d'une prestation en nature de l'assurance maladie à la déclaration de la situation familiale, ainsi qu'au lieu de résidence. Pour ce qui regarde la situation familiale, le lien n'est pas évident, l'éligibilité au remboursement des soins dépendant du seul état de santé et du statut de cotisant. Quant à la condition de résidence, également visée par l'amendement, elle est déjà satisfaite par l'article du code de la sécurité sociale qu'il vise. L'avis de la commission est également défavorable. Je veux juste rappeler que le bénéfice des prestations sociales est soumis à des obligations légales, notamment liées à la situation familiale et à la déclaration de la résidence en France. Le France. Le non-respect de l'une de ces conditions, par exemple l'absence de déclaration d'un changement de situation familiale ou d'un transfert de résidence à l'étranger, entraîne la suspension des prestations versées et la récupération des indus s'y rapportant. Lorsqu'un contrôle est effectué par un organisme de sécurité sociale, la personne doit bien justifier de sa situation ; à défaut, il est prévu la suspension des prestations.

Oh ! L'article R. 161-33-6 du code de la sécurité sociale oblige le titulaire de la carte d'assurance maladie à effectuer la mise à jour de sa carte en cas de changement de situation et au moins une fois par an à compter de la date d'émission de celle-ci. À cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition. Il existe donc bien un lien

afin d'unifier et de mettre en cohérence les pratiques sur l'ensemble du territoire, l'instruction générale relative à l'état civil créée en 1955 et utilisée par l'ensemble des officiers de l'état civil préconise l'utilisation généralisée d'un modèle d'acte de l'état civil. Il s'agit d'un modèle sous forme de rubriques afin de simplifier la tenue de l'état civil. Aujourd'hui, les mairies établissent les actes d'état civil sous ce format. En conséquence, un modèle unique d'acte d'état civil pourra être envisagé dans le cadre de la prochaine révision de l'instruction générale en question que le ministère de la justice compte mener. En ce qui concerne la lutte contre la fraude, l'uniformisation des modèles d'acte ne répond pas à votre objectif.

Cet amendement vise à rendre automatique la création du dossier pharmaceutique, sauf opposition de l'usager ou de son représentant légal, à l'instar de ce que les articles 45 et 50 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé prévoient du système de santé prévoient pour l'espace numérique de santé et le dossier médical partagé. La rédaction proposée est ainsi identique à celle prévue pour le dossier médical partagé. partagé. Or le dossier pharmaceutique abondera le dossier médical partagé. Cette proposition fait écho au rapport de la Cour des comptes pour 2020 publié le 25 février dernier présenté hier dans cet hémicycle, qui appelle de ses voeux la création automatique, sauf opposition du patient, du dossier pharmaceutique.

sont respectés et que ses données sont sécurisées conformément aux référentiels prévus. Hier, Mme la doyenne de la Cour des comptes nous a précisé

L'harmonisation des modalités de recueil du consentement entre le dossier médical partagé et le dossier pharmaceutique présenterait pour autre avantage d'améliorer la lisibilité de ces dispositifs pour les patients. Le titulaire de l'espace de santé se verra ainsi informé par le Conseil de l'ordre, préalablement à l'ouverture de son dossier, de la possibilité d'exercer son droit d'opposition avant que cette ouverture ne soit effective. Quel est l'avis de la commission spéciale La commission spéciale avait donné un avis défavorable à cet amendement, et je tiens à expliquer cette position en raison de sa contradiction apparente avec l'avis donné sur l'amendement n° 158 rectifié

En effet, l'article 9 de ce règlement, dont l'application est directe dans l'ordre juridique interne, prévoit que tout traitement de données personnelles de santé doit, pour exister, recueillir le consentement explicite du patient. Or le principe de l'ouverture automatique du dossier pharmaceutique substitue au consentement explicite un principe de consentement tacite du patient, ce qui paraît en contradiction manifeste avec le RGPD. Pour autant, la loi Santé a bien introduit cette substitution pour le cas du dossier médical partagé. Cependant, dans ce cas, la contradiction avec le RGPD n'est qu'apparente, puisque le consentement explicite du patient est préservé,

la plupart du temps par son médecin traitant à un moment où l'opposition du patient peut sans problème être recueillie. L'amendement de notre collègue Martine Berthet prévoit les mêmes précautions et assortit également le principe d'une ouverture automatique du dossier pharmaceutique de l'obligation de mettre le patient en situation d'exprimer son opposition préalablement à l'ouverture du dossier. il existe à mon sens une différence fondamentale avec le DMP : contrairement au médecin, le pharmacien ne sera pas à tout moment en mesure de recueillir cette opposition préalable, notamment lorsque le dossier pharmaceutique est créé par le pharmacien d'un établissement de santé ou lorsque la récupération de médicaments en officine se fait par une autre personne que le patient. La Cour des comptes a d'ailleurs soulevé ce problème dans son avis récent : « Il y a un déficit d'information des patients, qui ignorent souvent s'ils disposent ou non d'un dossier pharmaceutique. il existe donc un risque juridique important, auquel serait certainement exposé le pharmacien incité par la loi à créer automatiquement un dossier pharmaceutique, tout en n'ayant pas pu mettre le patient en situation d'exprimer son opposition préalable. C'est de cette inquiétude que la commission spéciale s'est fait l'écho, et non d'une réticence de principe au déploiement du dossier pharmaceutique, dont je saisis parfaitement les intérêts en termes de santé publique. Aussi, consciente des attentes de mes collègues en la matière, je sollicite, à titre personnel, l'avis du Gouvernement. Quel est C'est un avis favorable. Très bien ! Cet amendement vise à permettre la création automatique de dossiers pharmaceutiques, sauf opposition du patient. Ce passage de l'à l'est une recommandation du rapport de la Cour des comptes de février 2020- cela a été mentionné. Dans la lignée des évolutions relatives à l'espace numérique de santé et au dossier médical partagé, le Gouvernement est favorable à l'ouverture automatique du dossier personnel,

Outre cette mise en cohérence avec le régime d'alimentation à l'officine, une telle évolution simplifierait et fluidifierait le parcours de soins des patients entre la ville et l'hôpital. En effet, les admissions et les sorties de patients en établissement de santé constituent aujourd'hui des points de rupture dans leur parcours. Tout repose sur la capacité des patients à informer eux-mêmes les professionnels de santé les prenant en charge de leurs prises médicamenteuses en cours. Agrégeant les données pertinentes relatives aux patients, le dossier pharmaceutique permettrait de surmonter cette difficulté. Une telle évolution permettrait également de dynamiser l'intégration du dossier pharmaceutique au sein des systèmes informatiques hospitaliers, facilitant ainsi la consultation par les professionnels de santé à l'hôpital. Cette obligation entrerait en vigueur progressivement selon un calendrier fixé par voie réglementaire.

dans les hôpitaux -il se trouve que j'y ai travaillé voilà quinze ans -, l'initialisation de la partie prescription ne se fait pas au niveau du pharmacien. Je vous propose de retravailler cet amendement

Cet amendement a pour objet de simplifier les conditions d'exercice des biologistes médicaux en facilitant les modalités d'échange avec les prescripteurs afin d'éviter la réalisation d'actes inutiles. L'article L. 6211-8 du code de la santé publique permet au biologiste médical de réaliser des actes ne figurant pas sur la prescription, ou de ne pas réaliser tous les examens qui y figurent, lorsqu'il l'estime lorsqu'il l'estime approprié. Toutefois, la modification de la prescription ne peut être mise en oeuvre qu'après avoir été proposée au prescripteur, sauf en cas d'urgence ou d'indisponibilité. Par ailleurs, l'article L. 6211-9 du même code dispose que, lorsqu'il existe des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé, le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés avec ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur. Ainsi, ces deux dispositions supposent un échange préalable entre le biologiste médical et le prescripteur. Une discussion peut être complexe à engager, et la possibilité de modifier les prescriptions est très peu utilisée. Dès lors, il est proposé de mettre les articles L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique en cohérence et de faciliter la possibilité pour les biologistes médicaux d'ajuster les prescriptions au regard des recommandations scientifiques. Cette possibilité ne serait pas subordonnée à une validation par le prescripteur, même si ce dernier conserverait la possibilité de demander expressément sur l'ordonnance que la totalité des actes soit effectuée.

La législation actuelle permet à un médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques d'être coresponsable, lorsque la structure juridique du laboratoire de biologie médicale où il exerce autorise l'existence de plusieurs représentants légaux. aux termes de l'article L. 6223-5 du code de la santé publique, celui-ci ne semble pas pouvoir détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d'une société exploitant un un laboratoire de biologie médicale privé. Il est donc pertinent de clarifier le régime d'intégration des médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques au sein de ces structures et de reconnaître expressément l'existence de passerelles entre les deux professions.

Gouvernement ? Je partage votre souhait de coopération pluridisciplinaire. Sur ce point, de nombreuses avancées sont en cours. Cependant, de façon générale, je ne suis pas favorable à une modification de l'ordre de celle que vous proposez, c'est-à-dire touchant à la détention du capital de laboratoires de biologie médicale, sans débat approfondi avec les professions concernées. Le vecteur de l'amendement ne me semble pas apporter de garanties de méthode suffisantes pour une réforme touchant à l'outil de travail des biologistes. De plus, sur le fond, vous pointez du doigt une incohérence qui n'est qu'apparente, puisque, aujourd'hui, les spécialistes en anatomopathologie peuvent être désignés comme coresponsables d'un laboratoire de biologie médicale. Cela ne pose aucune difficulté. Enfin, on peut s'interroger sur le fait que cette avancée soit réservée aux anatomopathologistes,

Cet amendement vise à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'accréditation définitive des laboratoires de biologie médicale déjà accrédités pour au moins 50 % des examens de biologie médicale Compte tenu des efforts déjà consentis par les laboratoires en activité pour atteindre un haut niveau de qualité, nous souhaitons simplifier le processus d'accréditation de la totalité des examens en assouplissant le calendrier. Cet assouplissement permettra aux laboratoires d'achever le déploiement de leur stratégie d'accréditation au regard de leur périmètre d'activité au-delà du 1 novembre 2020. Il permettra également la bonne réalisation des évaluations nécessaires à l'accréditation du périmètre d'activité envisagé, sur la base des ressources d'évaluateurs disponibles.

assez contraint. La date du 31 octobre deviendrait celle du dépôt des dossiers d'accréditation auprès du Cofrac, et non la date d'accréditation elle-même. Le calendrier du processus d'accréditation reposerait alors sur le cycle d'accréditation de chaque laboratoire de biologie médicale.

par les pharmacies d'officine. Des difficultés persistent cependant dans des communes isolées ou peu peuplées, dans lesquelles les textes en vigueur ne permettent pas l'ouverture d'une officine, une population de 2 500 habitants étant requise.

2020, qui a été déclarée inconstitutionnelle pour des raisons de forme. Cette disposition prévoit que, dans le cas où la seule officine installée dans un village cesse son activité sans qu'un repreneur l'agence régionale de santé pourra autoriser la mise en place d'une antenne de pharmacie pour perpétuer l'accès à une offre pharmaceutique. Bien entendu, cette antenne sera rattachée à une pharmacie existante à proximité.

de l'article 34 afin de reprendre les termes exacts de la mesure adoptée par le Parlement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

d'un espace numérique de santé lui donnant accès à ses données de santé son dossier médical partagé et à différents services numériques référencés. Cet amendement vise à adapter ces dispositions afin d'assurer une meilleure convergence entre les deux outils que sont l'espace numérique de santé et le dossier médical partagé, apportant une clarification pour les usagers et une simplification pour les professionnels de santé, ainsi que les professionnels des secteurs médico-social et social. La création automatique, sauf opposition de la personne, est prévue au plus tard au 1 juillet 2021 pour le dossier médical partagé et au 1 janvier 2022 pour l'espace numérique de santé, alors que les deux outils sont profondément imbriqués et ont la même finalité. soit pour simplifier l'utilisation de l'espace numérique de santé ou pour rationaliser sa mise en oeuvre, il est apparu nécessaire de modifier la loi pour faire converger les dispositions relatives à l'ouverture de l'espace numérique de santé et du dossier médical partagé. Plus largement, l'espace numérique de santé doit être conçu comme un ensemble indissociable. L'usager n'aura plus à gérer qu'une seule identification, ainsi qu'un seul droit d'opposition pour l'ensemble. Afin de permettre la meilleure prise en charge possible du patient et de simplifier l'articulation entre le DMP et les autres outils de coordination, il est en outre essentiel d'ouvrir l'accès au DMP à l'ensemble des professionnels susceptibles d'intervenir dans sa prise en charge, notamment ceux du secteur médico-social. Cela vise à favoriser une homogénéisation entre les outils pour casser les silos entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social et simplifier l'articulation des systèmes d'information en santé. Une dernière modification tend à apporter une précision à l'article L. 1111-18 du code de la santé publique, afin que les règles d'accès au DMP s'articulent avec celles de l'espace numérique de santé à l'égard des services numériques référencés par les pouvoirs publics dans l'espace numérique de santé.

qui concentre en faveur du patient un ensemble d'applications de santé, et celle du dossier médical partagé. La mesure me paraît aller dans le bon sens. Ma position sur cet amendement diffère de celle que j'ai défendue sur le dossier pharmaceutique. En effet, les dispositions spécifiques du code de la santé publique prévoient que la personne ou son représentant légal est informé de l'ouverture de l'espace numérique de santé, ainsi que des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement, j'y insiste, à cette ouverture. ouverture. Cette application du principe de consentement tacite ménage tout de même, par cette obligation d'information préalable, la possibilité pour le patient d'exprimer une forme de consentement explicite,

article ... J'aimerais avoir confirmation de la part de Mme la secrétaire d'État que cet article vient résoudre une difficulté qui existe depuis les dernières réformes du code du sport en janvier 2016. Je

à une course à pied de 5 kilomètres organisée sous l'égide de la Fédération française d'athlétisme. Or il me semble que, s'il est apte à faire un ironman, il doit pouvoir faire 5 kilomètres en courant sans repasser devant son médecin

étions opposés au dispositif initial de l'article 37, qui visait à remplacer l'actuel certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive des mineurs par une déclaration de leurs parents en vue de l'obtention de la licence permettant l'inscription à une compétition. À l'appui de cette déclaration, les parents devaient remplir un questionnaire, et tout doute émanant des réponses aux questions entraînait alors une obligation de consultation d'un médecin avant l'obtention de la licence. Ce dispositif ne reposait ne reposait essentiellement que sur des déclarations non scientifiques, non médicales, et pas toujours éclairées des parents. Il posait donc un réel problème de responsabilité en cas d'accident Le texte issu d'un amendement de notre rapporteure ne nous satisfait pas davantage, malheureusement, car il pose d'autres problèmes. Il complète l'actuelle exigence de délivrance de certificat médical de non-contre-indication par le recours, « le cas échéant »-

Cette mention ne permet pas de connaître l'élément déclencheur de la consultation de prévention sanitaire et sociale obligatoire. Est-ce dans le cas d'une consultation faisant apparaître un doute sur la possibilité pour l'enfant de pratiquer un sport ou de participer à une compétition ? Est-ce dans le cas d'une impossibilité pour la famille de recourir à une consultation chez un praticien soit pour une raison financière, soit à cause d'un délai incompatible avec les exigences sportives ? Par ailleurs, les consultations obligatoires, dont les objectifs sont fixés par voie réglementaire, ne sont pas forcément réalisées par des médecins formés à détecter les troubles spécifiques de nature à interdire la pratique d'un sport donné. Dans ce contexte, et vu la complexité du sujet,

La mention « le cas échéant » vise à déclencher la consultation de prévention obligatoire lorsque le mineur n'a pas bénéficié de celle que prévoient les textes pour la tranche d'âge dans laquelle il se trouve.

éventuellement, faire des économies en évitant les cas dans lesquels un médecin serait sollicité deux fois plutôt qu'une. La commission spéciale ne peut donc être que défavorable à la suppression de cet article.

nous intégrerons dans le contenu type des consultations obligatoires la liste des questions à poser par le médecin traitant sur la pratique sportive et ses contre-indications. Enfin, il appartiendra aux parents, non pas de faire des déclarations fantaisistes ou littéraires, mais de remplir annuellement avec leur enfant un questionnaire relatif à la santé questionnaire relatif à la santé élaboré par le Haut Conseil de la santé publique, et qui contiendra des choses très basiques. Par exemple, une réponse positive à une question relative à un antécédent médical déclenchera

Aujourd'hui, l'obtention d'une licence sportive fédérale est subordonnée à la production d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins d'un an, quel que soit le type de pratique, loisir ou compétition, et quelle que soit la discipline. En théorie, les visites médicales liées à l'établissement de ces licences ne sont pas remboursables par l'assurance maladie, ce qui a trois conséquences : d'abord, un effet dissuasif pour les familles modestes et les familles nombreuses ; ensuite, l'existence indéniable d'un certain nombre de certificats de complaisance, bien qu'il soit difficile de chiffrer le phénomène ; enfin, le fait qu'en pratique les CPAM remboursent la majorité des consultations liées à l'établissement de ces certificats. Ce système, à l'utilité contestée dans son périmètre actuel, génère donc des dépenses sociales, un engorgement des cabinets médicaux à certaines périodes de l'année, notamment dans certaines zones sous-dotées en médecins généralistes, et une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs sportifs. Nous pensons qu'il serait judicieux de laisser la main aux fédérations sportives, conformément à l'article L. 231-5 du code du sport, lequel prévoit qu'elles « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires pour demander des certificats médicaux en fonction des pratiques et des niveaux de compétition. Le présent amendement vise donc à proposer une nouvelle écriture de l'article 37 pour permettre aux commissions médicales des fédérations sportives, dont l'existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts, le soin de fixer, par exception, lorsque cela apparaît justifié, les règles concernant l'obligation de présentation de ces certificats au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition. Il n'y aurait dès lors plus lieu de prévoir un régime distinct pour les mineurs ou pour les majeurs, ainsi que pour les disciplines à contraintes particulières. L'article 37 ainsi amendé

se posait alors la question de l'effectivité de la réponse à ce recensement. Le cliquet instauré a été le passage du permis de conduire, lequel était encore très désiré par les jeunes de cette génération.

délivrer du risque de voir cette démarche reconsidérée comme un avantage en nature par les Urssaf. Cette mesure est préconisée de longue date par les partenaires sociaux, par les représentants patronaux et par différents rapports, issus notamment du Conseil d'État. reprend également une annonce faite par le Premier ministre à l'occasion du comité interministériel pour les jeux Olympiques de 2024, le 4 novembre 2019. Il est donc urgent

n'est pas opposable. Il me semble pertinent, notamment dans le contexte de la préparation des jeux Olympiques de 2024, de favoriser le développement des activités sportives, qui sont de nature à améliorer la qualité de vie au travail. La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement. Cet amendement vise à exclure de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les « avantages fournis par l'employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ». Cette rédaction peut apparaître vague. Je rappellerai que, par principe, l'assiette des cotisations sociales doit intégrer l'ensemble des éléments de salaire et avantages en nature accordés par l'employeur. Néanmoins, dans le cadre actuel, il est déjà possible, sous conditions, de faire bénéficier ces salariés de tels avantages sans cotisations. Ainsi, les prestations en nature ou en espèces relatives à des activités sociales et culturelles servies par les comités d'entreprise sont exonérées de cotisations. La plupart des aides à l'activité sportive délivrées par le comité social et économique, ou par l'employeur en par l'employeur en l'absence de CSE, sont bien exonérées. En outre, afin de permettre le développement de la pratique du sport en entreprise, des travaux complémentaires sont en cours pour clarifier les critères d'exonération des avantages liés aux activités sportives, tels que la mise à disposition de locaux par les employeurs.

et à des conflits importants. Cette mesure favorisera le développement des sports et activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels. Aujourd'hui, le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air est entravé par une application stricte, à l'encontre des propriétaires et gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil. Sur ce fondement, par un jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la Fédération française de la montagne et de l'escalade, gestionnaire d'un site naturel pour le compte d'une commune,

Le tribunal a considéré que, quoique la fédération n'ait pas commis de faute, elle était gardienne de la chose à l'origine du dommage, en l'espèce le bloc de pierre qui s'était détaché. Cette décision a été confirmée en appel. Ce régime de responsabilité ne peut avoir pour effet que de freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l'accès à leurs terrains, ou à susciter,

Comme le souligne l'objet de l'amendement, le dispositif proposé favoriserait le développement des sports et des activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels. À ce titre, je tiens à souligner que ces propriétaires ou gestionnaires sont parfois des communes, ou d'autres collectivités territoriales.

La rédaction proposée vise seulement à limiter la responsabilité civile du gardien de l'espace et tend à supprimer une exonération jusqu'alors accordée par le code de l'environnement en matière de responsabilité administrative.

au profit d'un « document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ». L'état actuel du droit prévoit qu'un récépissé est délivré à toute personne admise à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Le récépissé autorise alors légalement cette personne à séjourner, mais aussi, le cas échéant, à voyager, à travailler ou à accéder aux droits sociaux. L'importance du document qu'il s'agit ici de remplacer est telle que, selon la Cimade, il est très fréquent qu'en raison de sa délivrance tardive ou de la remise d'une « attestation de dépôt » sans aucune valeur législative, des personnes perdent leur emploi, se voient demander des remboursements de trop-perçus par les caisses ou même soient interpellées et enfermées en centre de rétention administrative alors même qu'elles ont valablement introduit une demande et bénéficient selon la loi de tous leurs droits. Cette suppression de la référence législative aux récépissés est issue de la volonté du Gouvernement de déployer un nouveau service de dépôt en ligne et d'instruction dématérialisée des demandes de titre de séjour. Cela pose plusieurs problèmes. D'abord, le déploiement de la dématérialisation va à l'encontre de réels droits pour les étrangers, notamment les demandeurs d'asile, en état de grande précarité. Ces personnes éprouvent des difficultés à avoir accès à l'essentiel, et donc, bien évidemment à internet, sans parler des difficultés d'accès spécifiques de certains sites, ou encore de la barrière culturelle

Ensuite, au lieu de l'unique récépissé existant aujourd'hui, l'étude d'impact du projet annonce également la multiplication des types de documents provisoires- « attestation de dépôt de demande », « attestation de prolongation de l'instruction », « attestation de décision favorable » -, ce qui ne fera que rendre la procédure toujours plus complexe et illisible pour les usagers

peut simplifier l'accès des administrés à leurs droits. Toutefois, cette affirmation ne peut être généralisée à l'ensemble de nos concitoyens. Comme le rappelle le Défenseur des droits, l'objectif d'amélioration de l'accès aux droits ne sera pas atteint à marche forcée, sans tenir compte des difficultés bien réelles d'une partie de la population et des besoins spécifiques de certaines catégories d'usagers. surtout, si cette évolution conduit à une déresponsabilisation des pouvoirs publics en renvoyant aux associations ou au secteur privé la prise en charge de l'accompagnement de ces usagers qui serait nécessaire pour compenser les défaillances du service public. Cette dématérialisation peut aussi exclure ceux qui ne maîtrisent pas les outils informatiques : l'illectronisme concernerait 13 millions de Français, mais également des étrangers. D'ailleurs, notre groupe

n'est pas une solution magique à la saturation des guichets ; elle ne doit pas conduire à instituer des entraves à l'obtention de ces titres. Pour les personnes vulnérables, cette présence physique est essentielle, d'autant que l'obtention d'un récépissé en préfecture leur permet de rester sur le territoire le temps de l'instruction de la demande, de travailler et de séjourner à l'étranger. Il est donc important de préserver le caractère facultatif des démarches électroniques et de maintenir la possibilité de déposer une demande en préfecture et d'obtenir un récépissé.

échappera ensuite au législateur, alors qu'il s'agit d'une garantie essentielle pour l'exercice des droits du demandeur. Il n'est pas du tout acceptable

précisément la remise d'un récépissé à toute personne admise à soumettre une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Le récépissé est fabriqué par la préfecture et remis en main propre : c'est un document officiel sérieux.

encore plus remis en cause, car tout sera renvoyé à des décrets dont nous ne connaissons pas aujourd'hui la teneur. C'est donc à la fois une perte de droits pour les demandeurs et une perte de capacité du Parlement à garantir ces droits. Enfin, le contenu des futurs textes d'application est très flou.

L'article 38 clarifie les modalités de dépôt des demandes de titres de séjour. Il remplace les dispositions législatives prévoyant la délivrance de récépissés par une référence plus générale à des documents provisoires.

mais les ajustements proposés au présent article sont de portée très limitée. Il s'agit uniquement d'une clarification entre les dispositions relevant du domaine de la loi et celles qui

Le principe du droit temporaire au séjour pendant l'examen d'une demande reste évidemment affirmé au niveau législatif. Enfin, les auteurs de ces amendements redoutent les dangers de la dématérialisation envisagée par le Gouvernement.

Vous savez comme moi qu'on doit téléphoner pour prendre un rendez-vous, mais qu'on passe ensuite un certain temps, une partie de la journée,

Je ne peux pas répondre à la question de M. Leconte sur les documents sérieux : je ne connais pas de documents qui ne le soient pas. J'imagine que, quand on aura rempli sa demande,

est à M. Richard Yung. Cet amendement vise à garantir aux titulaires des documents provisoires dont on vient de parler le droit à l'exercice d'une activité professionnelle pendant la durée d'instruction de leur demande. C'est une demande qui est faite depuis de nombreuses années par les différentes associations qui suivent les demandeurs de titres de séjour ou d'asile,

ou pendant l'instruction de la demande sont actuellement prévus par l'article R. 311-6 du Ceseda. Ils sont en cohérence avec les droits attachés au titre de séjour, qui, eux, sont prévus par voie législative. La question de l'accès à

Il s'agit de rétablir au niveau législatif la possibilité pour ce public d'exercer une activité professionnelle, dans l'attente de la délivrance du titre, tout en renvoyant au niveau réglementaire le soin de matérialiser ce droit à travers la délivrance d'un document. Le Gouvernement partage l'intention de la rapporteure d'inscrire au niveau de la loi que les réfugiés et les titulaires de la protection subsidiaire bénéficient du droit d'exercer la profession de leur choix dans l'attente de la délivrance de leur titre de séjour.

sur les registres de l'état civil français ; c'est le tribunal de Nantes qui est spécialisé dans ces procédures. En outre, les Français dont le mariage a été célébré par une autorité étrangère ne sollicitent pas tous la transcription de leur acte de

que les modifications proposées n'entraîneraient pas une aggravation du risque de nullité et de fraude. C'est la raison pour laquelle la commission spéciale demande l'avis du Gouvernement émet un avis défavorable. Adopter les dispositions que vous proposez reviendrait à supprimer tout contrôle des mariages que les Français souhaitent contracter à l'étranger devant l'autorité locale compétente, tel que cela est effectué par les officiers d'état civil communaux lorsque le mariage est célébré en France. Or c'est dans l'optique d'apporter une protection identique aux Français souhaitant se marier à l'étranger que la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages a été adoptée. Il s'agit de s'assurer du consentement non vicié des futurs époux souhaitant contracter mariage, afin que cette institution ne soit pas détournée pour obtenir ou faire obtenir la nationalité ou d'autres objets. Ces dispositifs ont un sens et une utilité, puisque le parquet de Nantes a prononcé, en 2018, 365 oppositions à mariage ainsi que 93 oppositions à la transcription d'un mariage célébré à l'étranger.

Leconte. Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel la dématérialisation, contre laquelle nous n'avons rien, ne peut se faire au détriment des autres moyens de communication entre les autorités publiques et les citoyens, français comme étrangers. Si la dématérialisation

Cet amendement tend à consacrer dans la loi l'interdiction pour l'administration de communiquer uniquement sous forme dématérialisée. Cependant, la méthode proposée par cet amendement, transversal et de portée générale, ne me semble pas pas vraiment opérationnelle juridiquement. Son objectif est en partie satisfait par le droit en vigueur et son adoption introduirait de graves incohérences dans notre droit. La commission spéciale demande donc le

à l'issue de son expérimentation sans devoir passer par une modification législative. On peut aisément imaginer le fonctionnement de ce nouveau système : les candidats les mieux lotis, aussi bien financièrement que géographiquement, se verront rapidement attribuer une place pour passer l'examen ; les autres devront patienter, voire changer de département, pour pouvoir obtenir une place. Je rappelle la mise en garde de la commission spéciale dans son rapport : « Une éventuelle généralisation de la procédure d'inscription en ligne des candidats ne devra être réalisée qu'au regard de l'évaluation de l'expérimentation prévue, et uniquement si le bilan de celle-ci est est positif. » Nous nous étonnons donc que la commission spéciale ait adopté cet article sans modification. La situation est en effet assez cocasse : l'expérimentation en question d'une plateforme de réservation en ligne des places d'examen pratique dans cinq départements de la région Occitanie pour une durée de huit mois n'aurait été lancée qu'à compter du lundi 2 mars 2020 ! C'est ubuesque, mais, en matière de simplification, il est difficile de faire mieux, puisqu'il s'agit de tirer les conclusions d'une expérimentation quelques jours après sa mise en oeuvre. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 39. n° 92 rectifié. L'objectif affiché de la désintermédiation des places d'examen pratique du permis de conduire est de faciliter son accès aux nombreux candidats qui attendent des mois pour pouvoir se présenter. Or l'inscription directe en ligne encouragera le candidat à réaliser moins d'heures de conduite et à se présenter sans pour autant être prêt. L'article L. 221-1 A du code de la route prévoit que tout candidat se voit proposer une place d'examen sous réserve « d'avoir atteint le niveau requis L'inscription une plateforme risque d'accroître le nombre de candidats ajournés, qui devront se réinscrire, ce qui contribuera à allonger la liste d'attente et à déplacer le problème du sous-effectif d'inspecteurs. Elle interroge enfin sur la qualité de l'enseignement reçu en dehors des auto-écoles. La désintermédiation fait l'objet d'une expérimentation dans cinq départements de la région Occitanie. Il est d'ailleurs bien dommage que d'autres départements en plus forte tension, tels que ceux de l'Île-de-France, n'aient pas été inclus. Attendons donc l'évaluation de cette expérimentation avant de supprimer la base légale de la méthode nationale d'attribution en vigueur, qui a bien une valeur juridique. L'introduction de l'article L. 213-4-1 au sein du code de la route a « rendu nécessaire une modification de la méthode nationale d'attribution

de généraliser une disposition dont une loi précédente a décidé qu'elle ferait l'objet d'une expérimentation ! L'expérimentation a commencé avant-hier

À quoi sert-il de mettre en oeuvre une expérimentation si, avant même qu'elle ne commence, on décide de la généraliser ? Ce n'est alors plus une expérimentation, madame la secrétaire que la disposition que vous nous proposez est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2019, de laquelle toute généralisation d'un dispositif résultant d'une expérimentation nécessite au préalable une évaluation et la définition des conditions de son extension. Comme il n'y a pas d'expérimentation,

Or la commission spéciale considère que cette question relève du domaine réglementaire et non du domaine législatif. En effet, déterminer au niveau de la loi la méthode de répartition des places au permis de conduire crée une rigidité importante qui impose d'adopter une nouvelle loi à chaque fois qu'une modification est envisagée. Lors de l'examen du projet de loi Macron, le Sénat a supprimé l'article additionnel introduit par les députés qui entendait inscrire cette méthode dans la loi. Nous vous proposons d'être cohérents avec notre position d'alors

qui vient d'être lancée. Il n'y a donc pas de risque que cette méthode soit généralisée avant la fin de l'expérimentation, ce qui, au demeurant, n'aurait aucun sens. La commission spéciale

l'expérimentation a démarré, elle est en cours dans cinq départements depuis le 2 mars dernier et se poursuivra jusqu'au début de l'année prochaine. C'est sur cette base que nous préciserons les modalités

du code de la route, qui qualifie d'universel l'accès aux épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire et qui vise à garantir l'égal accès des candidats aux places d'examen du permis de conduire. De ce point de vue, une procédure numérique sera plus efficace que ce que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, vous

relèvent non du domaine de la loi, mais de celui du règlement. Nous pensons qu'elles relèvent de la loi lorsqu'elles définissent des principes généraux, comme c'est le cas à l'article L. 213-4-1 du code de la route, qui dispose que « la répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements ». En revanche, le second alinéa de l'article L. 213-4-1 du code de la route renvoie à des dispositions réglementaires la définition de la méthode d'attribution des places d'examen et des pièces nécessaires à l'inscription au permis de conduire. Selon l'avis du Conseil d'État, il n'est pas nécessaire d'introduire, dans les dispositions législatives, un renvoi à un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour définir les modalités d'attribution des places à l'examen du permis de conduire, un tel renvoi pouvant être prévu par les dispositions réglementaires. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer le second alinéa de l'article L. 213-4-1 du code de la route.

c'est bien le Conseil d'État qui nous a demandé de supprimer l'ensemble de l'article L. 213-4-1 que nous souhaitions initialement réécrire. Par ailleurs, comme je l'ai indiqué, l'article L. 221-1 A du code de la route

Symbole d'autonomie et passeport pour l'emploi, le permis de conduire rassemble, chaque année, plus d'un million de candidats. Depuis quelques années, le secteur de l'éducation routière s'est modernisé, notamment grâce aux avancées permises par le numérique et au développement d'offres en ligne. Ces offres ont contribué à améliorer le parcours de formation en permettant aux candidats qui souhaitent se former la liberté de choisir le parcours de formation qui leur convient le mieux. Le numérique a également apporté davantage de souplesse aux auto-écoles.

L'expérience montre d'ailleurs que la plupart des auto-écoles utilisent aujourd'hui ces logiciels en ligne, mais elles demeurent contraintes de faire venir les apprentis candidats dans leur local, quand bien même l'intégralité de l'évaluation se fait en ligne. Cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour tous les élèves de toutes les auto-écoles de réaliser cette évaluation initiale à distance. Cette modification du code de la route permettra aux auto-écoles de disposer de plus de flexibilité pour réaliser cette évaluation et d'optimiser l'usage des logiciels développés par la profession. cette évolution sera favorable au consommateur, qui bénéficiera de plus de souplesse pour comparer les offres des auto-écoles avant de s'engager. Cet amendement remet en cause la position d'équilibre proposée par la commission concernant le permis de conduire entre les acteurs traditionnels du secteur et les nouveaux entrants. De plus, d'après nos échanges avec les services du ministère, il serait susceptible de conduire à davantage de fraudes aux permis de conduire. L'avis est donc défavorable.

sur son parcours d'apprentissage prévisionnel. Elle n'est pas normée, comme peut l'être l'évaluation du code de la route, avec par exemple des réponses sur la signalisation qui seraient correctes ou incorrectes. Le contenu, qui varie selon les auto-écoles, présente des questions plus larges, comme l'expérience de la conduite des voitures, des motos, d'une bicyclette, la connaissance de la position des pédales ou de la boîte de vitesses, une première tentative d'évaluation de l'émotivité du candidat et sa capacité à retenir les indications du moniteur ou son sens de l'observation. Le niveau et les besoins de l'élève sont sans cesse réévalués au fur et à mesure de l'apprentissage. L'actuelle législation impose que l'évaluation ait lieu soit dans les locaux de l'auto-école, soit dans un véhicule dédié à l'apprentissage de la conduite, ce qui désavantage de manière évidente les auto-écoles en ligne et crée une inégalité face au droit. Or, aujourd'hui, un nombre croissant de candidats apprentis choisissent de s'inscrire au permis de conduire auprès d'une auto-école en ligne. en ligne. Libre à eux de faire ce choix. Il est assez paradoxal de leur demander, alors qu'ils se sont inscrits dans une auto-école en ligne, de réaliser cet examen de passage dans un lieu particulier ou dans une voiture, alors que l'objectif est simplement d'anticiper, de manière un peu théorique, la nature et le nombre d'heures que devra réaliser l'apprenti conducteur pour être au niveau du permis de conduire. L'amendement proposé vise à prendre en compte la situation de ces candidats et en conséquence à apporter une plus grande souplesse dans l'organisation de l'évaluation préalable, qui pourra, le cas échéant, se dérouler à distance un QCM, comme c'est du reste déjà parfois le cas des examens conduits par certaines écoles dans leurs locaux. La suppression des termes « dans le véhicule ou dans les locaux de l'établissement renforcera la sécurité juridique des contrats signés entre un apprenant et une école en ligne. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

Mme Jacky Deromedi. En matière d'assurance, en présence d'un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu'un sinistre survient, l'assureur mandate un expert afin d'évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l'assuré est en désaccord avec les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur, il dispose de la possibilité d'engager, à ses frais, une contre-expertise. Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue pourtant le principal outil de contestation de l'expertise des assurances, dont l'indépendance est parfois remise en question. Afin d'informer les assurés de l'existence de cette option, il convient de faire figurer, sur le contrat d'assurance, le possible recours à une contre-expertise, ainsi que le coût moyen de celle-ci. Quel est l'avis de la commission spéciale ? L'inscription d'une information relative à la faculté de réaliser une contre-expertise dans le contrat d'assurance soulève plusieurs problèmes. Tout d'abord, certains contrats d'assurance comprennent d'ores et déjà des clauses relatives à la prise en charge par l'assureur de telles prestations. Ensuite, l'information sur le coût moyen de la contre-expertise pourrait être très difficile à déterminer, puisqu'il dépend essentiellement du sinistre. L'information indiquée par l'assureur pourrait donc donner lieu à des contestations et ne serait, en pratique, que d'une faible utilité pour l'assuré. Enfin, le dispositif proposé ne comporte aucune condition d'application particulière. Il s'appliquerait donc aux contrats d'assurance en cours, qui devraient tous être modifiés sur ce point pour être en conformité avec la loi. Je sollicite donc le retrait de cet amendement Les modalités d'encadrement, d'évaluation des dommages en cas de sinistre, notamment la possibilité de recourir à une contre-expertise, relèvent normalement de la liberté contractuelle. Le Gouvernement est néanmoins conscient que des difficultés particulières peuvent parfois surgir, notamment en matière d'expertise en cas de catastrophe naturelle. naturelle. Il travaille à des mesures qui pourront être proposées dans le cadre de la réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Toutefois, à ce stade, il est trop tôt pour prendre une mesure sur le sujet, sans concertation préalable. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l'assuré par l'assureur de son droit de résiliation. Sans être encadré dans le temps, ce dispositif pourrait s'avérer doublement inefficace. D'une part, une information remise trop tard aurait pour conséquence de maintenir captif l'assuré pendant une année supplémentaire avant qu'il ne puisse faire jouer la concurrence. D'autre part, une information remise trop tôt n'inciterait pas l'assuré à effectuer les démarches nécessaires immédiatement, et celui-ci pourrait, faute de rappel ultérieur, ne plus s'en préoccuper. En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant la date choisie par l'assuréUne telle disposition permettrait à l'assuré d'être informé de l'approche de la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt dans un délai suffisamment restreint, lui offrant de manière effective l'information qui lui permettrait d'effectuer les démarches nécessaires à l'exercice de ses droits. Le recours à un délai encadré est courant. Celui-ci figure notamment à l'article L. 215-1 du code de la consommation depuis l'adoption de la loi Chatel du 28 janvier 2005. En outre, les établissements bancaires sont d'ores et déjà coutumiers de ce délai encadré. Celui-ci leur est imposé par exemple en matière de tarifs bancaires. Les assureurs n'y sont pas étrangers non plus. En effet, ceux-ci y sont soumis pour la majorité des autres contrats d'assurance. En outre, la mise en place d'un tel mécanisme dans le délai prévu par la proposition de loi ne pose assurément pas de difficultés. En 2005, le législateur avait laissé aux assureurs et à nombre d'autres professionnels un délai de six mois pour mettre en place le mécanisme qui serait instauré. Avec les progrès réalisés depuis, les établissements bancaires et les assureurs sauront se conformer aux mesures introduites dans un délai de quatre mois. Ainsi, l'instauration d'une telle disposition, d'ores et déjà mise en pratique pour d'autres types de contrats depuis de nombreuses années, permettrait de renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur. Quel est l'avis de la commission Le Sénat n'avait pas retenu un tel dispositif à l'occasion de l'examen de la proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur le 23 octobre 2019.

Même avis.

des termes du nouveau contrat d'assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré. En effet, lorsqu'un emprunteur souhaite changer l'assurance souscrite en garantie de son crédit immobilier, il présente un nouveau contrat au prêteur, qui doit en accepter ou en refuser les termes dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception. Or, en pratique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relève que certains établissements « ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d'assurance emprunteur ». Ainsi, l'emprunteur n'a en réalité pas d'autre choix que de conserver une assurance généralement plus chère. Ces procédés, qui visent à décourager les emprunteurs dans leurs démarches ou à différer la date de changement du contrat sollicité, sont rendus possibles par l'absence de sanction immédiate des prêteurs en cas de manoeuvres dilatoires. Par conséquent, l'instauration d'une acceptation tacite résoudrait cet écueil en imposant aux prêteurs d'accepter ou de refuser le nouveau contrat dans le délai imparti et rendrait véritablement effectif le droit au changement d'assurance emprunteur.

Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l'assuré par l'assureur de son droit de résiliation sur support papier ou tout autre support durable. Sans être encadré formellement, ce dispositif pourrait s'avérer inefficace. En effet, les pratiques des assureurs pourraient être divergentes et nuire à l'accessibilité de l'information pour les assurés. En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée sur l'avis d'échéance de l'assurance.

: La parole est à Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à s'assurer de la diligence des professionnels à appliquer la loi en remplaçant les sanctions administratives prévues par le texte par des sanctions pénales. Si la non-transmission de la fiche standardisée d'information fait l'objet de sanctions administratives, les établissements de crédit seront uniquement poursuivis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Or ces instances ne disposent pas de moyens humains suffisants pour pour traiter simultanément toutes les affaires dont elles sont saisies. À titre d'exemple, alors que son champ de compétences s'est élargi, notamment dans le cadre de la révision de la directive Services de paiement, a connu une baisse d'effectif de 6 % depuis l'année 2015. De ce fait, les sanctions administratives prévues par le présent article pourraient ne pas être appliquées. Il convient donc d'instituer des sanctions pénales. En conséquence, les actions en justice pourront être intentées par les victimes, les associations de consommateurs et les pouvoirs publics, dont la DGCCRF, qui dispose déjà du pouvoir de mettre fin aux mauvaises pratiques des « bancassureurs

avis. L'article 42 prévoit de dépénaliser les sanctions afin de garantir leur effectivité. C'est le fruit de nombreux échanges qui ont eu lieu au Sénat lors de l'examen de la proposition de loi déposée par le sénateur Martial Bourquin. Ces mesures avaient été adoptées à l'unanimité par le Sénat en octobre dernier.

Surtout, ce texte a été très sensiblement amélioré par notre commission spéciale pour faciliter la mise en place et la pérennité d'un tel dispositif pour les TPE. Le dispositif pourrait être ainsi maintenu au-delà des trois premières années de sa création, sans que les complexités propres à la négociation collective y fassent obstacle. Serait aussi pérennisé le dispositif de prime exceptionnelle créé par la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales de décembre 2018 et reconduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et serait supprimée la condition liée à l'existence d'un accord d'intéressement. En tant que membre de la délégation aux entreprises du Sénat, et au nom de notre collègue Élisabeth Lamure, qui préside cette dernière, nous pouvons nous réjouir de cette simplification, favorable à la fois aux chefs d'entreprise concernés et à leurs salariés. Enfin, nous prenons en compte les spécificités des TPE dans notre législation ! Je formule deux regrets cependant. Le premier tient au délai pourquoi ne pas avoir anticipé la situation des TPE, ce qui a freiné le versement d'une prime fin 2019, alors que l'on sait pertinemment qu'il leur est plus difficile d'appliquer une législation conçue pour des entreprises de plus grande taille ? Mon second regret tient à la modestie des dispositions de ce projet de loi en faveur de la simplification de la vie des entreprises. L'ambition affichée de développer l'activité et l'emploi dans nos territoires suppose de prendre en compte la réalité de la vie quotidienne, mais aussi des moyens des entreprises. Or qu'entendons-nous à l'occasion des nombreux déplacements de la délégation dans les territoires à la rencontre des ETI, PME et TPE ? Nous entendons des chefs d'entreprise courageux, responsables, qui sont étouffés par le poids de la réglementation, la défiance dont font preuve nombre d'administrations, l'instabilité juridique et fiscale ... Nous observons et nous nous inquiétons de l'absence persistante de traduction concrète, pour les entreprises, du discours sur « l'État au service d'une société de confiance », dont les dirigeants d'entreprises attendent toujours la concrétisation sur le terrain. Il faut donc avancer plus vite et plus loin, madame la secrétaire d'État, pour que le bon sens s'impose.

Vous avez supprimé le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés, contribuant au développement de l'épargne salariale, au détriment de l'augmentation du salaire brut. Or je rappelle que le salaire brut, c'est le salaire socialisé, le salaire socialisé, celui qui ouvre des droits à des prestations sociales, et donc une amélioration très faible du niveau de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Surtout, cette mesure est particulièrement coûteuse, puisque le Gouvernement a exonéré le forfait social sur ces contrats, entraînant un manque à gagner pour les caisses de la sécurité sociale de 660 millions d'euros pour 2020.

Vous voyez bien la différence ! C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Quel

rémunération complémentaire, qui représente d'ailleurs un pourcentage assez modeste de l'ensemble de la rémunération d'un salarié. Le Gouvernement ne se satisfait pas de la situation et souhaite que, d'ici à la fin du quinquennat, au moins 3 millions de salariés, dans les entreprises de moins de 250 personnes, puissent bénéficier d'un dispositif de partage de la valeur, contre 1,4 million aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'article 43 encourage les TPE à mettre en place un régime d'intéressement permettant de procéder par décision unilatérale de l'employeur lorsque c'est la première fois que l'intéressement est instauré dans l'entreprise. Les organisations Les organisations syndicales approuvent ce dispositif, précisément parce que les TPE ne sont pas organisées, en termes de dialogue social, comme des entreprises petites, moyennes ou grandes. Lorsqu'ils sont mis en place, ces dispositifs sont une source de motivation, de satisfaction pour les salariés au travail, en leur apportant un complément de salaire, mais surtout en leur donnant le sentiment de participer à une aventure commune, car l'entreprise est avant tout une aventure humaine collective. Ceux qui rencontrent des

Le Gouvernement propose de rétablir le texte initial dont vous avez été saisis. Il convient en effet de prévoir que le régime d'intéressement mis en place par décision unilatérale de l'employeur peut être reconduit par accord d'intéressement conclu avec les salariés ou leurs représentants. La mise en place unilatérale par l'employeur d'un dispositif d'intéressement est une dérogation au principe de la négociation d'un accord d'intéressement avec les salariés ou leurs représentants. Il s'agit d'une mesure d'amorçage destinée à faciliter la mise en place de l'intéressement dans les entreprises de moins de onze salariés dépourvues d'instances représentatives du personnel. Elle est limitée à une première mise en place de l'intéressement. À l'issue de cette première période d'application, l'employeur et les salariés auront pu s'approprier le dispositif, qui n'est pas si compliqué. La prolongation par voie négociée, par exemple la ratification d'un accord à la majorité des deux tiers des salariés, ne constituera plus, de notre point de vue, une difficulté. Cet amendement vise également à rétablir la condition d'existence ou de mise en place par l'entreprise d'un accord d'intéressement avant le 30 janvier 2020 pour pouvoir bénéficier de l'exonération sociale et fiscale prévue par l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 dans le cadre du versement de la prime exceptionnelle, y compris pour les entreprises de moins de onze salariés. Il s'agit en effet d'assurer dans la durée que les salariés bénéficieront d'une prime d'intéressement chaque année. Or, vous l'avez compris, la prime exceptionnelle est exceptionnelle Plusieurs mesures de simplification et d'accompagnement ont été prises pour faciliter la mise en place de ces accords, notamment dans les TPE. Les entreprises peuvent mettre en place un accord d'intéressement pour une durée inférieure à trois ans. Des modèles d'accord sont mis à disposition sur les sites ministériels. Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent directement mettre en oeuvre des accords d'intéressement négociés au niveau des branches professionnelles, ce qui leur permet de disposer d'un accord « clé en main » correspondant bien à l'activité sous-jacente de leur entreprise. En l'absence d'observation de l'administration, dans les six mois suivant leur dépôt, les accords d'intéressement sont intégralement sécurisés. Enfin, comme le prévoit le présent article, l'intéressement pourra être mis en place par décision unilatérale dans les entreprises de moins de onze salariés. Cette mesure est nécessaire à l'atteinte de notre objectif d'une meilleure diffusion des accords d'intéressement dans les petites entreprises, dans l'idée d'apporter à un peu plus de 1,5 million de salariés le bénéfice de ce supplément de rémunération.

par un accord d'entreprise ou un référendum. Cette limitation est apparue regrettable à la commission spéciale. En effet, s'il s'agit de lever un obstacle à la mise en oeuvre d'accords d'intéressement dans les entreprises qui sont trop petites pour organiser en leur sein un dialogue social formalisé, il n'est pas pertinent de limiter à une seule fois l'utilisation de cette facilité. Par ailleurs, Par ailleurs, même avec ces modalités simplifiées, la mise en oeuvre d'un dispositif d'intéressement peut représenter une formalité trop lourde dans certaines entreprises de très petite taille. Un substitut peut être le versement d'une prime.

Le texte adopté par la commission spéciale prévoit ainsi, pour les seules entreprises de moins de onze salariés, la pérennisation de ce dispositif et la suppression de la condition relative à l'existence d'un accord d'intéressement. La commission spéciale est donc défavorable

par le Gouvernement de développer l'intéressement dans les entreprises n'ayant pas les moyens ou la visibilité nécessaires pour mettre en place un dispositif d'intéressement en bonne et due forme. Or cet amendement tend à supprimer ces conditions pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Contrairement aux TPE, les entreprises plus grandes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs d'intéressement. Il me semble en outre qu'une pérennisation pour toutes les entreprises constituerait une niche fiscale et sociale dont il conviendrait d'évaluer les conséquences pour les finances sociales, notamment au vu des effets d'aubaine potentiels.

un système d'intéressement qui n'est pas juste une prime, mais qui repose aussi sur la définition de la réussite de l'entreprise ; ce ne sont pas uniquement des critères financiers.

Le présent amendement a pour objet de simplifier la procédure de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales au réseau des chambres de commerce et d'industrie, car le circuit de communication actuelle est lourd et provoque des retards. Actuellement, pour transmettre des données Actuellement, pour transmettre des données relatives à cette taxe, dont doivent être destinataires les chambres de commerce et d'industrie à des fins exclusives de réalisation d'études, la direction générale des finances publiques, détentrice des données, doit les communiquer à la direction générale des entreprises. Il appartient ensuite à cette dernière de les transmettre au réseau des chambres.

Le Gouvernement souhaite prolonger l'expérimentation de l'encadrement des promotions, afin de mieux réserver les effets économiques de ces dispositions, notamment sur les revenus des agriculteurs. Cet amendement tend à permettre de reconduire par voie d'ordonnance les dispositions de l'ordonnance du 12 décembre 2018 et de traiter la question plus complexe des conditions d'encadrement en volume des promotions. L'article 44 tel que modifié par la commission spéciale prévoit la prolongation pour quatorze mois seulement. Cette durée n'est pas suffisante du point de vue du Gouvernement. En effet,

des données sur les prix et, éventuellement, sur les industriels ; et encore : il faut attendre la publication des comptes des industriels et entrer dans une vision consolidée ! Mais ils n'auront pas nécessairement une analyse fine par région et par type de filière des agriculteurs. En tout cas, ils sont un peu inquiets quant à la disponibilité de ces données.

l'amendement proposé par le Gouvernement tend à rétablir, sous réserve de quelques ajustements mineurs, l'habilitation à légiférer par ordonnance supprimée par la commission spéciale. En premier lieu, le Sénat est par principe réservé sur le recours aux habilitations à légiférer par ordonnance. En second lieu, la prolongation proposée par l'habilitation à légiférer est particulièrement longue.

Par ailleurs, les aménagements envisagés par l'habilitation à légiférer ne sont pas expressément indiqués. La commission spéciale a donc substitué à l'habilitation à légiférer une prorogation sous conditions de certaines dispositions de l'ordonnance du 12 décembre 2018. D'une part, l'article résultant de nos travaux proroge de quatorze mois les dispositions précitées, ce qui correspond à une année d'application sur les principaux contrats agricoles, afin de disposer de plus de temps pour en mesurer les effets. D'autre part, l'article introduit dès à présent un correctif attendu des professionnels : la possibilité pour certains produits saisonniers de déroger à l'encadrement des avantages promotionnels en volume. Ce faisant, le dispositif adopté par la commission spéciale reprend la principale préconisation formulée par le rapport d'information sur l'application de la loi Égalim, remis au nom de la commission des affaires économiques du Sénat par nos collègues Daniel Gremillet, Michel Raison et Anne-Catherine Loisier. Cette disposition a par ailleurs été adoptée par le Sénat le 14 janvier dernier, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi modifiant la loi Égalim.

Le seuil de revente à perte ne constitue pas le point le plus contesté des dispositions de l'ordonnance issue de la loi Égalim de 2018. Les professionnels concentrent leurs critiques sur l'encadrement des avantages promotionnels. Dans ce contexte, les travaux précités du Sénat, tout comme d'ailleurs l'étude d'impact du présent projet de loi, insistent sur la nécessité de disposer de davantage de temps pour mesurer les effets du SRP sur les prix des denrées agricoles et sur les revenus des agriculteurs. C'est ce qui est important. C'est pourquoi la prorogation proposée par le

loi Égalim s'agissant particulièrement des produits saisonniers comme le foie gras. Le Gouvernement a été alerté par la filière palmipèdes avant la publication de l'ordonnance. Manifestement, il a été frappé de surdité.

le texte ASAP qu'il propose ne tient aucun compte des multiples interpellations de la filière et des travaux du Sénat. Ou peut-être est-il frappé de schizophrénie, au vu de l'étude d'impact, qui dresse exactement les mêmes constats Les faits sont têtus, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras communique les chiffres suivants : la filière a perdu 10 % des volumes vendus en 2019 ; les chiffres d'octobre et de novembre montrent des pertes de 35 % à 44 des volumes vendus en grandes et en moyennes surfaces. Les stocks résiduels suite aux méventes vont également provoquer une érosion des prix et réduire les volumes des productions à venir.

lourdement pour faire face aux mesures de biosécurité qui en avaient découlé, aidés en cela par l'État et les collectivités locales. Les discussions avec la grande distribution pour les contrats-cadres 2020 sont déjà achevées. La saison du foie gras se décide fin avril. Exclure la filière palmipèdes de l'encadrement promotionnel dès 2020 constitue un impératif. Des centaines d'exploitations, des ateliers artisanaux et des milliers d'emplois sont menacés. L'annonce de dérogations délivrées au cas par cas par la direction générale de la concurrence n'est ni satisfaisante ni juridiquement solide.

Cet amendement tend à ce que certaines informations issues de la déclaration sociale nominative soient transmises à l'Unédic, à France compétences et aux opérateurs de compétences. Les informations visées sont toutes celles qui ont trait à des sommes autres que des salaires, ainsi qu'aux prestations sociales versées par les organismes de protection sociale. Ce champ est potentiellement très vaste, et certaines de ces informations sont sans lien avec l'objet visé par les auteurs de l'amendement. En quoi l'Unédic, les OPCO ou France compétences auraient-ils besoin de connaître le détail des prestations sociales versées à chaque individu ?, l'amendement ne vise pas les salaires, qui constituent pourtant l'essentiel de la DSN. En outre, les informations contenues dans la DSN peuvent avoir un caractère personnel et sensible. Il ne me semble donc pas pertinent de multiplier les destinataires et les usages de ces informations. D'ailleurs, la mention des OPCO manque de précision. Tous les OPCO ou seulement celui qui est compétent pour l'entreprise à laquelle appartient le salarié ? Enfin, alors que la DSN constitue une rationalisation des flux d'information, prévoir une transmission à de multiples destinataires ne semble pas aller dans le sens de la simplification. La

La réception des données de la DSN est possible après formalisation auprès des services de l'État d'une expression du besoin pour exercer les missions attribuées par les textes en vigueur. Ces données sont ensuite intégrées à un arrêté qui fixe la liste des données transmises à chaque destinataire. En l'espèce,

tout individu qui exerce une activité lucrative sur la voie publique ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Le versement est de 150 euros sans utilisation d'un véhicule, majoré de 76 euros à 300 euros en fonction du nombre de véhicules utilisés. Il est délivré en contrepartie un récépissé de consignations qui doit être présenté à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats habilités. Le récépissé est valable trois mois. Le commerçant en question doit donc revenir tous les trois mois à la préfecture. l'exercice d'une activité commerciale impose dans toutes les situations de s'immatriculer auprès d'un centre de formalités des entreprises et de s'identifier auprès des administrations fiscale et sociale.

En outre, un indice public sur lequel les parties peuvent facilement se mettre d'accord existe pour chacune des matières premières concernées. Les parties n'auront ainsi qu'à définir dans leur clause le seuil de déclenchement et, éventuellement, les modalités d'activation de la clause.

la date d'entrée en vigueur. D'un point de vue économique, un tel mécanisme uniformiserait de manière très rigide le comportement des opérateurs, qui seraient privés de toute liberté pour moduler les répercussions des hausses des prix. Un fournisseur innovant ne pourrait pas profiter de ses gains de productivité pour absorber une hausse.

à moyen terme. Nous commençons à voir grâce à la loi Égalim des contrats sur cinq ans, notamment pour accompagner des signes d'amélioration de qualité. Cela permet d'amortir les investissements faits par les agriculteurs, avec une composante « prix du marché » et une composante

un guichet unique pour les subventions de l'État aux collectivités. Les communes, surtout lorsqu'elles sont petites et rurales, qui n'ont pas d'ingénierie hésitent souvent à demander des subventions, car la constitution des dossiers se révèle trop complexe et chronophage. Cet amendement tend à mettre en place un référent au sein d'une administration des services de l'État qui piloterait toutes les demandes de subventions et l'instruction des projets d'investissement. L'objectif est triple simplifier les procédures avec la constitution d'un seul dossier et ne plus demander, comme c'est le cas, les mêmes documents en plusieurs exemplaires ; accentuer le rôle de conseil de l'administration référente ; consommer des budgets qui, parfois, ne le sont pas, en ayant un réel rôle de coordinateur entre les différents partenaires financiers.

En outre, le Gouvernement continue de prendre des mesures fortes pour l'accompagnement des communes, notamment rurales, dans leurs demandes de subventions et la simplification de leurs démarches. La plupart des dotations de soutien à l'investissement local font ainsi l'objet, depuis 2019, d'une instruction interministérielle unique, afin de mieux assurer l'accès des collectivités territoriales à l'information recherchée.

Pour ce qui concerne le droit des marchés publics, en effet, les CPI sont les conseils qui interviennent le plus en amont auprès des entreprises pour protéger et valoriser leurs innovations, essentielles à leur développement. Si l'on en restait

Dans le cadre des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, les avocats et les CPI sont amenés à travailler ensemble au sein d'une même structure, dans le respect des mêmes obligations déontologiques. proposée est donc nécessaire. Elle va également dans le sens d'une meilleure valorisation de l'innovation sous toutes ses formes, celle-ci constituant indéniablement le véritable levier de croissance pour nos économies européennes.

par le second. Quel est l'avis de la commission spéciale ? La finalité de cet amendement est compréhensible : il s'agit de faciliter l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle en calquant les obligations qui lui sont applicables en matière de secret professionnel sur celles qui s'appliquent aux avocats.

Il est de jurisprudence constante que, lorsqu'un avocat échange avec un autre professionnel pour le compte d'un client commun, et même si ce professionnel est soumis à son propre secret professionnel, cela n'a pas pour effet de faire bénéficier leur échange de la confidentialité et de la protection offertes par le secret professionnel des avocats. Cette règle revêt une importance particulière en matière d'enquête, puisque les correspondances échangées entre un avocat et ces professionnels peuvent être saisies chez le client comme chez l'avocat sans que puisse être invoqué le secret professionnel. Le présent amendement vise à remettre en cause cette règle au seul profit des conseils en propriété industrielle, et notamment des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice. Or rien ne justifie une telle dérogation, d'autant que les conseils en propriété industrielle ne sont pas les seuls à pouvoir constituer de telles sociétés avec les avocats. Les textes relatifs à l'interprofessionnalité visent également les experts-comptables ou les officiers publics et ministériels. En tout état de cause, une telle modification nécessiterait une véritable analyse de son impact, en particulier sur la mise en oeuvre des pouvoirs d'enquête des autorités judiciaires ou administratives. Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable

des dispositions positives pour l'information des maires en matière d'implantation d'éoliennes,

Il est malheureusement d'autres dispositions avec lesquelles nous sommes en désaccord : la suppression de la Commission de suivi de la détention provisoire, du Conseil national de l'aide aux victimes et de la Commission nationale d'évaluation des politiques de

environnementale, le remplacement de l'enquête publique par une consultation, dans des conditions qui nous paraissent contestables, l'ouverture de la possibilité d'exécuter certains travaux